L'ordre du jour appelle l'examen de trois projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l'approbation de conventions internationales. Pour ces trois projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d'examen simplifié. Je vais donc les mettre successivement aux voix.

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification de la Convention n° 190 de l'Organisation internationale du travail relative à l'élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail

2019, réunie à l'occasion de sa cent huitième session, dite session du centenaire, la conférence générale de l'Organisation internationale du travail (OIT) a adopté la convention n° 190 visant à éliminer la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Cette convention, nous le savons, était particulièrement attendue par les États membres de l'OIT, nos concitoyens, les organisations non gouvernementales (ONG) ou encore les partenaires sociaux. Le 23 juillet dernier, l'Assemblée nationale a su répondre à ces attentes en adoptant en première lecture le projet de loi qui vous est présenté aujourd'hui. C'est donc solennellement que j'appelle votre chambre à voter en faveur de ce texte pionnier et protecteur des droits des femmes au travail, qui établit la première norme contraignante, de portée universelle, pour éradiquer la violence et le harcèlement dans le monde du travail. L'ambition de la convention est d'assurer à chacun et à chacune d'entre nous le droit d'évoluer dans un monde du travail où aucune violence ne peut avoir sa place. Cette ambition se traduit par un article unique, qui vise à ratifier la convention n° 190 de l'OIT, elle-même composée d'un préambule et de vingt articles. L'article 1 de cette convention introduit la première définition internationale de la violence et du harcèlement au travail, qui sont « un un ensemble de comportements et de pratiques inacceptables, [ ...] qui ont pour but de causer [ ...] un dommage d'ordre physique, psychologique, sexuel ou économique, en comprenant la violence et le harcèlement fondés sur le genre la violence et le harcèlement au travail sont protéiformes. Il nous faut viser l'ensemble de ces actes inacceptables, encore trop souvent passés sous silence et subis dans la sphère professionnelle. Cette convention vient ainsi reconnaître le droit de chaque personne à vivre dans un monde du travail libéré de la violence et du harcèlement. C'est un droit essentiel, mesdames, messieurs les sénateurs, et c'est une véritable avancée que de le reconnaître. Cette convention porte une attention particulière aux violences fondées sur le genre. À ce titre, l'article 2 rappelle que personne ne saurait être victime de la violence et du harcèlement au travail. Ainsi, le texte impose aux États l'ayant ratifié des obligations de moyens pour protéger chacun dans le monde du travail, et ce quel que soit son statut : salarié, contractuel, stagiaire, bénévole, demandeur d'emploi, Il s'agit de ne laisser personne de côté, sans protection particulière. La convention est complétée par la recommandation n° 206, qui n'est pas un texte contraignant soumis à la ratification des États, mais qui vient en préciser la mise en oeuvre. Il était essentiel Il était essentiel de définir un niveau de normes qui garantisse les protections fondamentales contre le harcèlement et les violences et qui, dans le même temps, puisse être adopté par le plus grand nombre de pays. Le champ Le champ d'application de la convention est particulièrement large. Il doit être lu à la lumière d'obligations qui sont, quant à elles, adaptées aux responsabilités de chacun. La convention prévoit ainsi que les employeurs doivent prendre des « mesures appropriées correspondant à leur degré de contrôle » pour prévenir la violence et le harcèlement dans le monde du travail, dans la mesure où cela est « pratiquement « pratiquement réalisable tous les moyens dont ils disposent pour lutter contre les violences et le harcèlement. En se faisant le porte-parole de l'Union européenne et de ses États membres durant les deux années de négociation, la France a joué un rôle moteur dans la discussion comme dans l'adoption de ce texte. Mesdames, messieurs les sénateurs, le résultat est à la hauteur de nos attentes. Vous l'aurez compris, le présent projet de loi revêt une importance majeure pour notre pays qui, grâce- je l'espère -à votre approbation, sera parmi les premiers à ratifier ce texte ambitieux. de la convention viendra consacrer l'engagement du chef de l'État en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Dès le début du quinquennat, le Président de la République a en effet pris un engagement solennel et très fort, en faisant de l'égalité entre les femmes et les hommes la « grande cause nationale » du quinquennat, dont la lutte contre le harcèlement et les violences dans le monde du travail fait pleinement partie. Quatre ans après, le constat est sans équivoque : les actes ont suivi les paroles et les engagements que nous avions pris. Cela s'est traduit par la tenue du Grenelle des violences conjugales, destiné à lutter plus efficacement contre les violences faites aux femmes, notamment dans le monde du travail.

Toujours très concrètement, nous avons intégré les violences conjugales dans le guide relatif à l'égalité professionnelle à destination des TPE-PME pour accompagner ces petites entreprises dans la prise en charge de ces situations de violence. Enfin, le futur plan Santé au travail (PST 4) abordera cet enjeu dans son volet relatif à la qualité de vie au travail, afin de renforcer la mobilisation de tous, y compris celle des entreprises, dans la lutte contre ces violences.

De manière plus globale, la responsabilité de l'employeur en matière de harcèlement et de lutte contre les violences est extrêmement bien établie dans les textes, conformément à l'obligation qui lui est faite de veiller à la santé et la sécurité de ses salariés. Nous avons également créé dans la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel un référent en matière de harcèlement sexuel dans toutes les entreprises de plus de 250 salariés, afin de prévenir, d'agir et de lutter contre les agissements sexistes et les faits de harcèlement sexuel au travail. Le Gouvernement, par la voix de la ministre du travail Élisabeth Borne, a encore récemment rappelé sa détermination à ratifier la convention n° 190, à l'occasion du Forum Génération Égalité, qui s'est tenu à Paris le 2 juillet dernier, en présence d'une soixantaine de chefs d'État et de gouvernement, ainsi que d'acteurs du monde entier.

Tous ensemble, agissons dès maintenant et donnons-nous tous les moyens possibles pour éradiquer les violences et le harcèlement sous toutes leurs formes Avec la ratification de cette convention de l'OIT, compatible avec notre droit interne, tous les dispositifs de protection que nous avons mis en place sont aujourd'hui réunis pour faire de la France un pays moteur et exemplaire dans la prévention et la répression de la violence et du harcèlement Les partenaires sociaux ont également un rôle actif à jouer en matière de lutte contre le harcèlement et les violences au travail, en application des obligations de négociation qui leur incombent, à l'échelon tant des entreprises que des branches. Ils ont aussi un rôle à jouer pour négocier des dispositifs ambitieux qui n'ont pas tous vocation à relever de la loi. Je pense notamment à la question de la prise en compte des violences conjugales dans l'organisation du travail au sein de l'entreprise.

Il est sans doute souhaitable d'aller plus loin dans ce domaine, mais cela suppose d'abord une concertation entre les partenaires sociaux. Vous connaissez mon attachement au dialogue social. Ce sont là des sujets extrêmement délicats, car ils sont à l'interface entre vie personnelle et professionnelle,

et de la traduire en mesures concrètes, adaptées aux réalités des défis auxquels nous faisons face dans le monde du travail. une fois ratifiée, les principes qu'elle fixe devront être appliqués, afin que l'ensemble des acteurs du monde du travail puissent se l'approprier. Mesdames, messieurs les sénateurs, tel est l'enjeu du présent projet de loi, qui doit permettre à la France de continuer à se montrer exemplaire en ratifiant la première ce texte visant à éradiquer la violence et le harcèlement au travail. La parole

l'intense action du Gouvernement -, la lutte contre la violence et le harcèlement au travail a été inscrite à l'ordre du jour de la Conférence internationale du travail dès 2015. Trois ans plus tard, la campagne #MeToo et plusieurs affaires judiciaires très médiatisées ont rappelé l'importance et l'urgence de légiférer sur le sujet, afin d'enrayer ce fléau, dont les femmes payent, ici comme ailleurs, un lourd tribut. Il est d'ailleurs intéressant de relever qu'aucune étude statistique fiable n'existe sur les violences sexistes et sexuelles au travail, ce qui tend à démontrer que le phénomène est insuffisamment pris en compte, voire tabou, y compris en France. C'est pourquoi l'Organisation internationale du travail s'attelle, à juste titre, à élaborer des normes statistiques internationales. « C'est dans ce contexte que l'Organisation internationale du travail a adopté, au mois 2019, à une très large majorité, la convention n° 190, qui constitue la première norme internationale dans ce domaine. Sa portée est historique et son contenu est à la hauteur de l'enjeu : toutes les personnes que j'ai auditionnées se sont félicitées des avancées qu'elle comporte, et ont salué le rôle moteur joué par le Gouvernement à l'occasion des deux sessions de négociation. « Toutefois, les organisations syndicales, comme les ONG, regrettent que les mesures les plus ambitieuses aient été intégrées à la recommandation n° 206, qui n'a aucune portée normative et qui, par conséquent, n'est pas soumise à l'examen du Parlement.

Je ne peux que regretter un tel choix, car l'examen du texte nous offrait l'occasion d'avancer sur le sujet en droit national, en complément des mesures gouvernementales mises en place à la suite du Grenelle des violences conjugales, entre autres.

Ce nombre est insuffisant pour les entreprises qui comptent plusieurs milliers de salariés et qui sont présentes sur plusieurs sites. Par ailleurs, ces référents ont souvent d'autres prérogatives, ce qui limite le temps qu'ils peuvent consacrer à cette mission. « Aucun moyen, par exemple un local pour recevoir les victimes qui les saisissent, ne leur est alloué, et certains référents ne bénéficient d'aucune formation adéquate. D'après les syndicats, certains référents abandonneraient leur fonction, faute de pouvoir l'exercer correctement. proposition est d'améliorer la formation et la vigilance à l'égard des violences et du harcèlement dans le milieu professionnel. Lors du Grenelle des violences conjugales, les experts ont souligné certaines lacunes en matière de formation et se sont prononcés en faveur d'une amélioration du dispositif, à destination de tous les professionnels en contact avec les femmes victimes de violences, comme les cadres intermédiaires et supérieurs et les personnels des ressources humaines. « En outre, et c'est ma troisième proposition, dans une économie mondialisée, le devoir de vigilance des entreprises doit s'étendre à l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement, afin de veiller au respect des dispositions de la convention, y compris par les sous-traitants et les fournisseurs. « J'en viens maintenant à la prise en compte des violences domestiques dans la sphère professionnelle.

les organisations patronales semblent hostiles à cette idée, préférant une stricte séparation des sphères privée et professionnelle. Ces deux sphères sont pourtant intimement liées ! « Comment peut-on imaginer qu'une femme victime de violences conjugales puisse en faire abstraction une fois arrivée sur son lieu de travail ? Comment peut-elle occuper au mieux son poste de travail si elle ne trouve aucune aide pour se reconstruire ? Je considère à cet égard que le lieu de travail doit aussi être un lieu d'écoute, d'accueil et d'accompagnement des victimes. Il y va d'ailleurs de l'intérêt de l'entreprise elle-même. « J'appelle donc le Gouvernement à créer les conditions d'un tel accord, en invitant les partenaires sociaux à débattre de cette question dans le cadre du quatrième plan Santé au travail, en cours d'élaboration. Pour ce faire, le PST 4 devra prévoir un volet spécifiquement consacré aux violences et au harcèlement pour que des discussions tripartites puissent avoir lieu. Il s'agit là de ma quatrième proposition. de grandes entreprises françaises ont une politique volontariste pour faire reculer les violences dont leurs collaboratrices peuvent être victimes, y compris lorsqu'il s'agit de violences domestiques. Ces actions sont généralement le fait de grands groupes qui disposent des ressources nécessaires à leur mise en oeuvre, et les progrès enregistrés sont bien souvent le fruit de négociations entre les partenaires sociaux. Aussi me semble-t-il important d'intégrer cette thématique aux négociations annuelles sur la qualité de vie au travail, obligatoires dans les entreprises dotées d'organisations syndicales représentatives. C'est l'objet de ma cinquième proposition. J'observe qu'en matière de prise en compte des violences faites aux femmes la France accuse un certain retard par rapport à des pays comme l'Espagne, le Canada ou la Nouvelle-Zélande. Dans ces pays, les victimes peuvent bénéficier d'un aménagement de poste et d'horaires,

vise à garantir l'autonomie économique des victimes de violences- vous y avez déjà fait référence, monsieur le secrétaire d'État. « Lorsqu'elles démissionnent, ces victimes peuvent désormais bénéficier des allocations chômage et débloquer leur épargne salariale, laquelle n'existe cependant pas dans toutes les entreprises. Même si elles sont bienvenues, ces mesures se révèlent insuffisantes pour garantir aux victimes une indépendance économique leur permettant de s'éloigner d'un conjoint violent. En effet, la perte d'un emploi, qu'elle soit consécutive à une démission ou à un licenciement, précarise les victimes de violences conjugales et obère leur indépendance économique. C'est pourquoi il est primordial de protéger les victimes de violences domestiques contre le licenciement. le 1 janvier prochain, la France prendra la présidence du Conseil de l'Union européenne. À ce titre, notre pays devra jouer un rôle moteur pour, d'une part, que les États membres ratifient et appliquent les dispositions de la convention dans des délais raisonnables et, d'autre part, que la lutte contre la violence et le harcèlement au travail constitue l'une des priorités de cette présidence. Nous devons montrer l'exemple et faire progresser notre droit interne pour que la convention soit appliquée de manière ambitieuse et que la violence et le harcèlement en milieu professionnel reculent enfin. Notre commission a adopté à l'unanimité ce projet de loi, preuve que ce sujet nous concerne tous et qu'il dépasse les clivages politiques. J'espère que le Gouvernement entendra mon appel à aller plus loin. » La parole est à M.

nous ayons ce débat sur la ratification de la convention n° 190 de l'Organisation internationale du travail sur le harcèlement et les violences dans le monde du travail. Le débat nous permet de mettre en lumière la tendance de ce gouvernement à prendre, dans les grandes enceintes multilatérales, par ailleurs louables, mais que l'on peine ensuite à retrouver dans les politiques menées dans notre pays. Cette convention en est un excellent exemple. L'omniprésence des violences et du harcèlement dans le monde du travail, liés ou non au genre, est aujourd'hui une réalité incontestable. Je rappellerai les chiffres que nous connaissons toutes et tous : en 2019, 30 % des femmes salariées en France ont déjà été harcelées ou agressées sexuellement sur leur lieu de travail, et 70 % d'entre elles n'en ont jamais parlé à leur employeur. Comment s'en étonner lorsque l'on sait que dénoncer ces faits a fréquemment des conséquences négatives pour elles ? Si les femmes sont significativement plus touchées, n'oublions pas que d'autres groupes y sont aussi très exposés, notamment les travailleurs et les travailleuses précaires, dont le secteur domestique. À ce sujet, nous sommes ébahis que la France n'ait pas encore souhaité ratifier la convention n° 189, cohérente avec la présente convention n° 190. Il était donc urgent d'élaborer une telle convention. Nous constatons avec satisfaction qu'elle permet d'englober de nombreuses formes de violences et de harcèlement, compréhension large du monde du travail. Elle permettrait, par exemple, de mieux protéger les aides familiales, ces membres d'une famille travaillant sans statut salarié, dont 71 % disent avoir été victimes d'atteintes sexistes. telle ratification ne serait pourtant qu'une demi-victoire si nous ne tenions pas compte de la recommandation n° 206, qui y est associée. C'est apparemment le projet du Gouvernement, qui considère que notre législation y est déjà conforme, bien que celle-ci ne permette pas, par exemple, de contraindre les entreprises à agir dans le domaine des violences domestiques. Malgré les alertes des ONG, des syndicats ou des organes consultatifs, rien n'y fait le Gouvernement n'a pas l'intention de mettre notre législation en conformité avec ses nouvelles obligations vis-à-vis de la convention, celle-là même qu'il a grandement contribué à faire adopter. Monsieur le secrétaire d'État, nous vous invitons à remédier à ces incohérences en vous appuyant notamment sur l'étude d'impact de la CGT et de deux ONG, droits de l'homme (CNCDH) du 28 avril 2020, ainsi que sur le rapport de la commission des affaires étrangères. Il faut déposer rapidement un texte prévoyant les nouvelles mesures qui s'imposent désormais. Parmi ces mesures, il sera indispensable de mieux protéger les victimes, notamment en améliorant la formation des cadres et en reconnaissant les atteintes comme des accidents du travail.

de la démission à une perte involontaire d'emploi lorsqu'elle est motivée par des faits de violence ou de harcèlement. La France, riche d'une longue histoire en matière de protection des travailleurs et, dans une certaine mesure, des travailleuses, a joué un rôle crucial faire aboutir cette convention, participant à consacrer enfin le droit « de toute personne à un monde du travail exempt de violence et de harcèlement, y compris de violence et de harcèlement fondés sur le genre

Il n'est pas inutile de rappeler ici qu'une travailleuse sur trois a déjà été victime de harcèlement sexuel au travail. Nous ne sommes donc pas face à un phénomène mineur, et il est plus que temps d'agir pour ne pas banaliser ni minimiser ces violences. Il faut également rappeler que, malgré leur obligation de protection des salariés, 82 % des employeurs n'ont, à l'heure actuelle, rédigé aucun plan de prévention contre les violences sexuelles et sexistes. Il n'est donc pas étonnant que la grande majorité des victimes ne se sentent pas en confiance pour alerter les directions concernées,

de mars 2020, j'avais interrogé la ministre du travail de l'époque pour que le processus soit lancé. Il y avait en effet urgence. D'une part, cette convention n° 190 s'attaque pour la première fois à une problématique malheureusement structurante et omniprésente dans nos sociétés. D'autre part, par sa portée normative internationale,

Si la convention et, surtout, la recommandation qui l'accompagne sont ambitieuses, et si la France a joué un rôle important au sein de l'OIT, je dois néanmoins regretter, comme bon nombre d'associations et d'organisations syndicales, que le Gouvernement considère que son adoption puisse se faire à droit constant. En ce sens, je partage les recommandations de Mme le rapporteur Nicole Duranton pour aller plus loin. Il n'est pas possible, monsieur le secrétaire d'État, de considérer que notre droit actuel suffit à atteindre les objectifs affichés. En rester là serait véritablement une occasion manquée. Comment peut-on estimer que la législation actuelle est suffisante et satisfaisante quand on sait, par exemple, que les « référents harcèlement », créés en 2018, ne sont absolument pas formés et ne disposent d'aucun moyen pour exercer leur mandat ? Comment peut-on considérer que notre droit suffit, quand on sait que les violences et le harcèlement ne font pas partie des thèmes obligatoires des négociations annuelles sur la qualité de vie au travail ? De plus, comment ne pas regretter que, pour l'instant, les employeurs- et rien ne les y oblige ! -refusent très majoritairement de

outre, pourquoi ne pas vouloir inscrire dans notre droit l'interdiction des licenciements de victimes de violences conjugales ? Quant aux violences exercées au travail, il nous faut également avancer sur la voie d'une facilitation des procédures d'éloignement des victimes et des harceleurs. Les nombreuses propositions en ce sens devraient être mises en oeuvre renforcement des droits à congé spécifique, aménagements de poste, possibilité de percevoir des allocations chômage pour les victimes qui démissionnent, dispense de préavis de départ, etc. Au-delà, il convient également de s'interroger sur la baisse continue du nombre des inspecteurs et des inspectrices du travail, malgré les alertes des syndicats et celles de la Cour des comptes. Faut-il rappeler ici que l'article 4 de la convention impose impose bien aux États signataires, dont la France, de garantir des moyens d'inspection et d'enquête efficaces pour les cas de violence et de harcèlement ? Ce n'est pas la seule incohérence de ce gouvernement, bien aidé, il faut le dire, par ses prédécesseurs. Je citerai la création du comité social et économique (CSE), en remplacement des anciennes instances paritaires, qui a conduit à une dilution des problématiques, rendant plus difficile l'élaboration de plans thématiques. La ratification de la convention constitue un premier pas non négligeable. Notre groupe la soutiendra, en appelant de ses voeux à ce qu'elle ne soit pas appliquée, mais au contraire, qu'elle soit pleinement l'occasion

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, l'émergence du mouvement #MeToo, ces dernières années, nous rappelle la persistance du harcèlement et de la violence dans nos sociétés, particulièrement à l'égard des femmes. Le monde du travail n'est bien sûr pas épargné. En 2014, le Défenseur des droits publiait une enquête selon laquelle une femme sur cinq avait déjà été victime de harcèlement sexuel sur son lieu de travail. le manque d'études statistiques fiables sur les violences sexistes et sexuelles au travail démontre que le sujet est trop peu pris en compte, voire sous-estimé.

Cette égalité doit s'exercer partout, et notamment dans le monde du travail. La ratification de la convention n° 190 de l'Organisation internationale du travail relative à l'élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail va va dans ce sens. Cette convention est la première norme internationale sur la violence et le harcèlement qui s'exerce « à l'occasion, en lien avec ou du fait du travail ». Elle prévoit l'instauration de moyens de protection et de prévention, et souligne la nécessité de garantir des voies de recours et de réparation. Elle incite également les États membres de l'OIT à mettre en place des orientations, des formations et des actions de sensibilisation dans ce domaine. La France sera le neuvième pays à ratifier cette convention, ce dont nous nous réjouissons. Dans le cadre de la délégation aux droits des femmes, nous avons pu échanger sur ce sujet avec de nombreuses structures, des organisations syndicales, des représentants de l'Organisation internationale du travail ou encore des membres du Gouvernement. Tous ont salué l'implication du Gouvernement français dans les négociations. D'après l'étude d'impact du présent projet de loi, la législation française est conforme aux articles de la convention : il n'est donc pas nécessaire de changer nos règles pour ratifier et appliquer cet accord. Toutefois, un collectif d'associations et d'ONG, que la délégation aux droits des femmes a auditionnées au mois de juin dernier, conteste cette interprétation juridique. Elles recommandent de faire évoluer la loi sur plusieurs points, notamment renforcer les moyens et les prérogatives des référents harcèlement, obliger les employeurs à agir en matière de violences domestiques, et mieux tenir compte de la situation des victimes de violences. De tels dispositifs s'appliquent déjà en Espagne, au Canada ou encore en Nouvelle-Zélande. La ratification de la présente convention aurait pu permettre une véritable réflexion au niveau national.

contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Si cette convention doit nous interroger à l'échelon national, la réflexion doit également être La France prendra la présidence du Conseil de l'Union européenne à partir du 1 janvier 2022. À ce titre, elle doit jouer un rôle moteur pour que les États membres ratifient, puis appliquent les dispositions de cette convention.

aux violences à caractère sexiste, de bousculer les stéréotypes sexistes, de combler les écarts entre les hommes et les femmes sur le marché du travail et de parvenir à une participation égale dans les différents secteurs de l'économie. Pour davantage d'efficacité, il semble nécessaire d'uniformiser les différents dispositifs de lutte contre les violences faites aux femmes et de faire front commun. Je souhaite à cet égard saluer la démarche de ma collègue Nathalie Goulet, qui a pris l'initiative de déposer une proposition de résolution européenne, que j'ai d'ailleurs cosignée, qui vise à mettre en place une base juridique commune pour lutter contre les violences fondées sur le genre.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, après deux ans de négociations, la convention n° 190 de l'Organisation internationale du travail relative à l'élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail a été approuvée. C'est bien entendu un progrès fondamental pour la condition des travailleurs.

d'un texte qui reflète les valeurs républicaines d'humanisme et d'égalité qui nous sont chères. Tout le monde doit pouvoir accéder aux mêmes droits au travail, le premier d'entre eux étant de pouvoir exercer sereinement son activité, sans pression, qu'elle soit physique ou psychologique. Notre collègue François Patriat l'a rappelé : il s'agit d'une préoccupation récente à l'échelle internationale, qui suit cependant, dans beaucoup de pays, des mouvements de revendication très anciens.

le quotidien de millions de femmes dans le monde sur leur lieu de travail. Le mouvement #MeToo a indéniablement fait avancer les choses, mais beaucoup reste à faire. Cette question touche tous les pays, les moins comme les plus développés. Aux États-Unis, d'un tiers des travailleurs américains estiment avoir été victimes de conduites abusives au travail pendant leur vie. Toutefois, il va de soi que dans les États institutionnellement fragiles, l'appréhension des phénomènes de harcèlement est plus difficile. En ma qualité de corapporteur spécial de la mission « Aide publique au développement », je rappelle l'existence de politiques visant à lutter contre les mauvaises pratiques au travail. L'aide au développement du syndicalisme est un exemple de levier d'action.

nous devons aussi nous interroger sur notre législation : est-elle à la hauteur des enjeux ? Notre pays apparaît comme un bon élève. Cependant, les acteurs de la société civile nous demandent, à juste titre, de faire davantage. Mon groupe, le RDSE, est bien naturellement favorable à toutes les démarches qui vont dans le sens d'un renforcement de la lutte contre le harcèlement au travail. Plus globalement, nous sommes vigilants sur la condition des salariés au travail, sous tous ses aspects. Mon collègue Christian Bilhac l'a rappelé lors de l'examen, en juillet dernier, de la proposition de loi sur la santé au travail, dont le rapporteur Stéphane Artano est également très sensible à ces questions. Aussi, nous approuverons ce projet de loi, qui ouvre la voie à une meilleure prise en compte des violences exercées à l'égard des personnes vulnérables. Nous resterons toutefois attentifs aux suites concrètes qui lui seront données.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la convention que nous examinons est la première norme internationale sur la violence et le harcèlement qui s'exercent « à l'occasion, en lien avec ou du fait du travail Afficher, au niveau international, la volonté de protéger les salariés, mais beaucoup plus largement les apprentis, les stagiaires, les demandeurs d'emploi et les bénévoles, qui plus est, avec une vigilance renforcée

n'existait aucun instrument international consacré à la lutte contre les violences et le harcèlement au travail. Aucune définition n'avait été proposée pour couvrir l'ensemble des actes de violence ou de harcèlement. Aujourd'hui, nous posons des mots sur des actes inacceptables, et nous adoptons une définition universelle, qui s'appliquera à chaque État membre de l'OIT, en tout cas à tous ceux qui adopteront cette convention. La convention n° 190 qui est soumise à notre ratification incite les 187 États membres de l'OIT à mettre en place des actions de formation et de sensibilisation ou des orientations pour protéger les salariés contre toutes les formes de violence et de harcèlement. Il est demandé aux États signataires de prévoir des dispositifs de protection et de prévention, ainsi que des voies de recours pour obtenir réparation. que tout est parfait. Seulement, la recommandation n° 206, qui complète la convention et précise les modalités de sa mise en oeuvre, n'a aucune portée normative.

Lors de cette conférence annuelle, les délégués des gouvernements, des travailleurs et des employeurs des 187 États membres de l'OIT ont déclaré viser le même objectif : éliminer la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Notre groupe votera évidemment en faveur de cette première norme internationale sur la violence et le harcèlement qui s'exercent « à l'occasion, en lien avec ou du fait du travail Comme le précise notre collègue Nicole Duranton dans son rapport, les organisations syndicales et les ONG auditionnées ont toutes salué l'engagement du Gouvernement lors de ces négociations. Elles ont notamment souligné que la France avait pleinement assumé le rôle de porte-parole du bloc européen, et avait ainsi largement contribué à la création d'un instrument international de portée ambitieuse. Nous pouvons nous en féliciter.

Tout le monde est concerné : les travailleurs et tous les autres acteurs du monde du travail, à savoir les salariés, les employeurs, les apprentis, mais aussi les stagiaires, les demandeurs d'emploi et les bénévoles. Le texte couvre tous les secteurs : le public comme le privé, les secteurs relevant de l'économie formelle ou informelle.

« respecter, promouvoir et réaliser le droit de toute personne à un monde du travail exempt de violence et de harcèlement », ainsi que les « principes et droits fondamentaux au travail », à adopter une législation et des politiques garantissant « le droit à l'égalité et à la non-discrimination dans l'emploi et la profession La convention détaille ensuite les mesures de protection et de prévention à mettre en oeuvre, puis le contrôle de leur application et, enfin, l'importance des actions de formation et de sensibilisation.

Notre rapporteur, Nicole Duranton, formule un certain nombre de propositions : tout d'abord, renforcer les prérogatives et les moyens des référents harcèlement après avoir dressé un bilan ; améliorer la vigilance en imposant, par exemple, aux cadres intermédiaires et supérieurs, ainsi qu'aux personnels des ressources humaines, une obligation de formation sur le thème de la violence et du harcèlement au travail- il est aussi proposé d'inclure un volet consacré à la violence et au harcèlement dans le prochain plan Santé au travail

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, si « le travail éloigne de nous trois grands maux » comme l'écrivait Voltaire, il est parfois malheureusement un lieu de violence ou de harcèlement. l'Organisation internationale du travail a adopté une convention qui entend renforcer la lutte contre ces violences. Nous soutenons pleinement cet objectif. La première des nécessités est de dresser un état des lieux, afin de connaître l'ampleur de ces phénomènes, les mécanismes à l'oeuvre et les personnes qui en sont victimes. Nous devons avoir une idée précise du problème si nous voulons y apporter une réponse adéquate. L'adoption de cette convention nous incite à nous doter d'outils statistiques qui permettront d'acquérir ces connaissances. Pour éliminer les angles morts, tous les acteurs du monde du travail devront également être à même d'identifier les faits de violences et de harcèlement. Les victimes de ces pratiques sont souvent des personnes vulnérables ; il nous faut veiller à les en protéger. Nous devrons également nous assurer que notre arsenal juridique, et notamment pénal, nous permettra de lutter efficacement contre ces pratiques. Leurs auteurs doivent être fermement condamnés. Cette convention, à elle seule, ne suffira pas à éliminer la violence au travail. Elle constitue la première étape d'une évolution qu'il nous faudra poursuivre. Les différentes auditions menées par notre rapporteur, Nicole Duranton, dont je salue ici le travail,

quant au fait que les dispositions les plus ambitieuses ont été reléguées dans le texte de la recommandation n° 206, qui est, elle, dépourvue de toute valeur normative. Nous comprenons ces regrets, mais nous savons aussi que la modération est souvent le prix du consensus, lequel contribue au progrès. Il nous semble en outre que la modération est la conséquence de la prudence, qui nous commande de ne pas agir brutalement contre une menace qui reste aujourd'hui mal identifiée. Nous sommes également conscients que cette convention devra trouver sa place dans l'ordre normatif français, alors que l'Union européenne exerce sur ce sujet une compétence concurrente à la nôtre. Nous sommes pleinement favorables à ce que le Gouvernement se coordonne avec les autorités européennes, afin que ces dispositions soient mises en oeuvre le plus efficacement possible. Les problématiques du harcèlement et de la violence au travail nous concernent tous. Au sein de cet hémicycle, nous avons le devoir de lutter contre ces pratiques.

Nous ne pouvons que saluer son adoption à l'unanimité, la semaine dernière, par la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. La lutte contre le harcèlement et la violence dans le monde du travail est un sujet grave, qui mérite que les instances internationales, telles que l'OIT, s'en saisissent. Il faut se féliciter que la France ait porté, dès 2015, cette question à l'ordre du jour de la Conférence internationale du travail qui se réunit tous les ans à Genève. Il aura fallu deux ans de négociations avec les autres États membres de l'OIT pour que cette convention soit adoptée à une large majorité. Mes chers collègues, la convention marque un tournant, puisqu'il s'agit du premier instrument juridique international consacré à la lutte contre le harcèlement et la violence dans le monde du travail. C'est inédit et cela démontre une réelle prise de conscience sur ces sujets importants, alors même que la définition et la répression de ces infractions diffèrent selon les pays. nous devons nous féliciter de la manière dont sont rédigés les articles 1 à 3, qui définissent les deux notions et leur champ d'application. La définition du harcèlement est volontairement large, ce qui permet de couvrir les différents cas de harcèlement et de violences au travail, dont le cadre juridique varie d'un État à l'autre. Concernant les champs d'application, il convient de souligner qu'eux aussi sont larges. En effet, toutes les catégories de travailleurs sont mentionnées,

Il importe que la convention soit applicable à cette nouvelle ère du travail en distanciel, dans laquelle, nous le savons, les frontières entre la sphère privée et la sphère professionnelle sont de plus en plus poreuses. Sur ce point, l'article 3 est suffisamment explicite, puisque la convention vise les actes « s'exerçant à l'occasion, en lien avec ou du fait du travail ». Cela signifie que les temps de repos, les logements de fonction, les déplacements professionnels et la communication sont pris en compte. J'en viens maintenant aux conséquences concrètes pour les États signataires de cette convention qui, contrairement à ce qui a pu être dit, sont soumis à de réelles obligations. C'est l'objet des articles 4 à 6 et des articles 7 à 9. Dans un premier temps, ces États devront « promouvoir et réaliser le droit de toute personne à un monde du travail exempt de violence et de harcèlement

et des politiques garantissant le droit à l'égalité et à la non-discrimination dans l'emploi et la profession ». Enfin, ils devront mettre en place des mesures de prévention et prévoir des garanties pour l'exercice des droits de recours et de réparation pour les victimes. En ratifiant cette convention, les États s'engagent non seulement à agir concrètement contre les violences et le harcèlement au travail, mais aussi à rendre compte de leur action auprès de l'OIT dans ce domaine, deux ans après

Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, vous l'aurez compris, le groupe Les Républicains votera en faveur de la ratification de cette convention.

le projet de loi qui vous est soumis aujourd'hui vise à ratifier l'accord signé à Bruxelles le 27 janvier 2021 par la France et dix-huit États membres de la zone euro, puis par l'Estonie le 8 février 2021, portant révision du traité instituant le Mécanisme européen de stabilité (MES). Cette révision s'inscrit pleinement dans le projet d'approfondissement de l'Union économique et monétaire, auquel une nouvelle impulsion a été donnée par le Président de la République lors de son discours de la Sorbonne le 26 septembre 2017. Quatre ans plus tard, des avancées significatives ont été enregistrées en ce qui concerne la mise en oeuvre de ce programme ambitieux grâce au patient travail de conviction et aux intenses efforts de négociation du Président de la République et du Gouvernement français auprès des institutions et de nos partenaires européens. Nous ne comptons pas nous arrêter là, car il reste encore beaucoup à faire, mais force est de constater que les fondations d'une zone euro plus résiliente, plus intégrée et plus solidaire sont désormais posées. Parmi les avancées concrètes en vue de l'approfondissement de l'Union économique et monétaire, on peut citer le mécanisme de soutien aux dépenses de chômage partiel dans les États membres, dit SURE, rapidement mis en place en mai 2020, et le dispositif d'endettement conjoint Next Generation EU, destiné à financer des investissements et les réformes dans les États membres pour soutenir la relance.

celle de renforcer et de compléter le deuxième pilier de l'Union bancaire, à savoir le mécanisme de résolution unique (MRU), dont l'objectif est de veiller à ce que les défaillances bancaires soient gérées efficacement et soient le moins coûteuses possible pour les finances publiques. Le traité révisé institue en effet un dispositif de soutien, dit, sous la forme d'une ligne de crédit du MES au Conseil de résolution unique (CRU), l'agence européenne chargée de la résolution bancaire. Cet outil précieux complétera les ressources déjà disponibles au sein du Fonds de résolution unique (FRU) et renforcera la crédibilité des institutions dans la gestion des crises financières. Le FRU a été créé dans le cadre de l'Union bancaire en 2014. Il est alimenté par les contributions des secteurs bancaires des États participants jusqu'à ce qu'il atteigne son niveau cible minimal, soit 1 % des dépôts bancaires en 2024. Ces ressources sont mobilisables sous certaines conditions dans le cas où la mise à contribution des actionnaires et des créanciers ne serait pas suffisante pour prendre en charge la totalité du coût de la résolution d'une banque en difficulté.

Pour rembourser ce prêt, le CRU lèvera des contributions sur les banques de l'Union bancaire, si bien que celui-ci sera,, neutre budgétairement pour le MES et pour ses actionnaires- les États membres de la zone euro.

Par ailleurs, cette réforme porte également sur les missions plus traditionnelles du MES, celles qui concernent l'assistance financière aux États membres de la zone euro. Elle vise à rendre plus efficaces et plus attractifs les instruments dits « de précaution » pour les États dont les fondamentaux économiques sont sains, mais qui ont besoin d'une aide ciblée et ponctuelle pour surmonter une difficulté passagère ou un choc limité et, ainsi, échapper à la mise en place d'un programme d'ajustement macroéconomique complet, si la crise devenait plus sérieuse. Concrètement, pour avoir accès à l'un des deux instruments de précaution du MES, l'État en question n'aura plus besoin de signer un protocole d'accord comprenant des engagements contraignants sur la mise en oeuvre de réformes structurelles, mais seulement une lettre d'intention dans laquelle il s'engagera à respecter, à tout moment, les conditions associées à l'utilisation de la ligne de crédit de précaution. En outre, la réforme clarifie le mandat et le rôle du MES à l'égard de la Commission européenne dans le cadre de la préparation, de la mise en oeuvre et du suivi des programmes d'assistance financière.

Ainsi, grâce au nouveau traité, un petit groupe minoritaire de détenteurs obligataires ne pourra plus prendre en otage une restructuration de dette dans l'espoir d'obtenir un meilleur traitement pour lui-même. Le Gouvernement reste pleinement mobilisé pour poursuivre les travaux visant à achever l'Union économique et monétaire, notamment sa composante bancaire, l'Union bancaire, pour que les bénéfices attendus se matérialisent, y compris en termes d'intégration. La parole

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous examinons ce matin le projet de loi autorisant la ratification de l'accord modifiant le traité instituant le Mécanisme européen de stabilité (MES), le Sénat étant la première assemblée saisie. Il comprend un article unique visant à autoriser la France à ratifier cet accord modificatif. L'accord en question a été signé en janvier dernier par la France et les dix-huit autres États membres de la zone euro. L'objectif est de faire en sorte que ces dispositions s'appliquent dès le début de l'année prochaine, ce qui pourrait toutefois être plus difficile que prévu. Pour mémoire, le MES a vu le jour en octobre 2012 sous la forme d'un traité intergouvernemental conclu entre les seuls États membres de la zone euro. Il présente donc la particularité d'être en dehors de l'ordre juridique de l'Union européenne. Le MES vise à mobiliser des ressources financières et à apporter un soutien à la stabilité économique et financière de la zone euro. Il a pris le relais des programmes mis en place dans l'urgence lors de la crise de la zone euro. Mes chers collègues, il me semble important de répondre à trois questions principales. Tout d'abord, pourquoi modifier le traité initial ? Ensuite, quelles sont les modifications opérées ? Enfin, quelle analyse pouvons-nous en faire ? Commençons par le contexte et l'objectif de l'accord modificatif. Devant la crise de la zone euro, deux principales réponses ont été apportées. La première réponse est intervenue

De ce point de vue, avec une capacité totale de 500 milliards d'euros de prêt, le MES a pleinement rempli son rôle. Depuis sa création, il a porté assistance à trois pays- la Grèce, l'Espagne et Chypre -pour un montant total de 89 milliards d'euros.

Si les deux premiers sont effectifs depuis 2015, la garantie européenne des dépôts reste à finaliser pour passer d'une harmonisation des cadres juridiques nationaux à un véritable système européen.

D'autre part, le cadre actuel de l'Union bancaire ne préserve pas parfaitement les finances publiques des États en cas d'entrée en résolution d'une banque. La résolution d'une banque repose en effet sur trois éléments un renflouement interne, un renflouement externe par l'intermédiaire du Fonds de résolution unique, dont les ressources sont issues des contributions du secteur bancaire et, éventuellement, un soutien de l'État membre concerné. C'est la motivation principale ayant conduit à l'accord modificatif : concrétiser pleinement l'objectif initial de rendre étanches les dettes souveraines et le secteur bancaire. L'ambition initiale était de transformer le MES en un fonds monétaire européen. Une telle évolution aurait permis de l'intégrer dans l'ordre juridique européen, d'unifier les rôles du MES et de la Commission européenne et, surtout, de compléter les ressources du FRU par un filet de sécurité. Aucun compromis n'a toutefois été trouvé parmi les États membres, ce qui a rapidement conduit à recentrer l'ambition sur une modification du MES. C'est l'objet de l'accord modificatif dont le projet de loi vise à autoriser la ratification.

d'éviter que le contribuable d'un État membre soit mis à contribution pour venir au secours d'une banque en difficulté. C'est mieux ! Pour cela, il est proposé de permettre au MES de prêter jusqu'à 68 milliards d'euros au CRU par le biais d'une ligne de crédit renouvelable. Le filet de sécurité peut être appréhendé comme une sorte de prêt relais du MES au CRU, le temps que le secteur bancaire rembourse les montants qui lui ont été versés pour le soutenir. Mes chers collègues, vous pourriez être tentés de me dire que nous transférons la charge d'un contribuable d'un État membre vers les banques de la zone euro. En schématisant, le filet de sécurité reporterait la charge du contribuable grec sur les banques françaises. Dans ces conditions, quel intérêt le présente-t-il ? En réponse, laissez-moi vous indiquer que la procédure actuelle ne cantonne pas la charge éventuelle au seul contribuable grec, mais implique tous les États membres. pour aider une banque en difficulté, un État membre peut bénéficier d'un prêt du MES. Soyons clairs : l'évolution proposée ne conduit pas à davantage de mutualisation, mais fait remonter l'aide à la résolution d'un cran, en transférant la charge du contribuable au secteur bancaire. Il s'agit donc bien de la concrétisation d'un principe posé dès 2012. Pour autant, ne soyons pas naïfs

Le premier concerne l'entrée en vigueur du filet de sécurité. L'objectif affiché est volontariste, puisque les États parties ont souhaité avancer sa création au 1 janvier 2022. Cependant, le processus de ratification prend du temps : un recours a été formé en Allemagne, et plusieurs pays n'ont pas encore présenté d'instrument de ratification.

S'il vient doubler les capacités du FRU, l'ensemble pourrait ne pas suffire, selon la banque mise en résolution. S'agit-il selon vous d'un risque réel,

relaie une inquiétude des banques françaises sur la façon dont celles-ci pourraient être mises à contribution en cas d'utilisation du filet de sécurité. Elles souhaitent que le CRU

Pouvez-vous, monsieur le secrétaire d'État, nous assurer que la France plaidera en ce sens et limitera ainsi au strict nécessaire l'éventuelle contribution de nos banques en cas de recours au filet de sécurité ?

Loin de prôner l'entraide entre les États ayant l'euro pour partage et de les aider ainsi à sortir du joug des marchés financiers, il s'est révélé être une réponse inadaptée aux constats posés à la suite de la crise financière et bancaire de 2008. Les modifications introduites par l'accord qui nous est soumis n'y changeront rien : les marchés financiers seront les grands bénéficiaires de ce texte, loin des ambitions du discours de la Sorbonne du Président de la République. La création du filet de sécurité vient entériner l'impuissance du Fonds de résolution unique, abondé par les banques elles-mêmes pour pallier une crise bancaire. Ainsi, 75 milliards d'euros sont attendus pour 2024, soit 1 % des dépôts bancaires couverts- c'est largement insuffisant. Dans ce cadre, les États membres devraient engager leurs finances publiques, des prêts, pour sauver les banques qui s'adonnent à des pratiques spéculatives et trop souvent déraisonnables. « Cela ne coûtera rien aux États membres », a-t-on entendu en commission. Peut-être, mais aucune modalité de remboursement par les banques n'est prévue dans cet accord. On abondera donc le CRU de 68 milliards d'euros sans savoir comment on les récupérera ; on négociera une fois la crise venue, dans l'urgence, avec l'éternel dogme mis en avant par les ministres européens les banques sont « » ! Eh oui ! Elles ont droit à l'aléa moral, au soutien public. De plus, l'argument de la neutralité budgétaire risque de s'effondrer devant une crise systémique financière et bancaire, d'autant que les mesures prudentielles ne sauraient être suffisantes pour l'éviter.

Le prétendu assouplissement d'un nouvel instrument d'assistance financière de précaution est un leurre. La suppression du mémorandum, document d'engagement à des réformes structurelles, n'y changera rien.

Voyez donc la faiblesse de cet argument pour le moins paradoxal. La France ne pourrait pas bénéficier de cette procédure prétendument plus souple et moins stigmatisante, même dans sa forme allégée par le présent accord, car l'état de nos finances publiques ne permet pas de remplir

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l'Union européenne fait régulièrement l'objet de controverses et de débats : atteinte à la souveraineté ou monstre technocratique pour certains, chantre d'une orthodoxie budgétaire dépassée pour d'autres, union des peuples et garantie d'une paix durable pour d'autres encore. Le projet européen repose résolument sur l'idée de coopération et de solidarité. De la constitution d'un marché commun à la création de la zone euro, la monnaie demeure sans aucun doute le fil rouge de ces dernières décennies. Entre crises successives et renforcement de l'intégration économique, financière, puis bancaire, les États membres de la zone euro ont toujours été enclins à faire muter les tenants et les aboutissants de la zone monétaire européenne. Si ces évolutions ont pu être tardives, poussives, parfois contre-productives, les échanges et les débats n'ont jamais cessé. Et le projet de loi autorisant la ratification de l'accord modifiant le traité instituant le Mécanisme européen de stabilité,

Le Mécanisme européen de stabilité est un fonds commun de créances pour pallier la défaillance d'un État membre. Les ressources mobilisées par ce dispositif doivent permettre de faire face aux obligations financières. Parallèlement à la mise en place progressive des différents piliers de l'Union bancaire sous l'empire du droit européen, le Mécanisme européen de stabilité, fondé sur un traité intergouvernemental, offre une complémentarité essentielle aux outils préexistants. Héritier du Fonds européen de stabilité financière (FESF) et du Mécanisme européen de stabilisation financière (MESF), le MES fait l'objet de velléités de révision depuis plusieurs années. Finalisé le 4 décembre 2019 par l'Eurogroupe, révisant le traité a été signé par les dix-neuf États membres de la zone euro les 27 janvier et 8 février 2021, conjointement avec l'accord modifiant l'accord intergouvernemental sur le transfert et la mutualisation des contributions au Fonds de résolution unique. unique. Les modifications du traité, qui nous sont soumises aujourd'hui au titre de l'article 53 de la Constitution, reposent sur quatre évolutions principales qui ont déjà été largement évoquées : faciliter les restructurations des dettes souveraines ; renforcer le rôle du directeur du MES et l'indépendance du mécanisme ; réviser les instruments de précaution ; et, bien sûr, créer un filet de sécurité. Ces évolutions visent à renforcer la résilience de la zone euro face aux crises à venir.

l'accord modifié précise le fonctionnement de la facilité de soutien du MES au Conseil de résolution unique (CRU). Dans un premier temps, le conseil des gouverneurs approuve d'un commun accord l'octroi de la facilité- une ligne de crédit de dix ans renouvelables -sur demande du CRU. Dans un second temps, le conseil d'administration du MES décide de l'octroi des prêts et des versements jusqu'à 68 milliards d'euros. Cet article décrit également la procédure d'urgence qui peut être activée en cas de menace et abaisse le seuil d'approbation des prêts et versements à 85 % des voix exprimées en conseil d'administration. Il s'agit donc bien, dans des circonstances extrêmes, de simplifier le recours au filet de sécurité, en évitant qu'une poignée d'États puisse en bloquer le fonctionnement. Pour rappel, l'Allemagne, la France et l'Italie détiennent respectivement 21 %, 16 % et 14 % des droits de vote.

La distance géographique et politique entre le quotidien des Français et les actions de l'Union européenne ne doit pas être ignorée. L'information et la pédagogie, surtout sur un texte aussi complexe, doivent doivent faciliter la compréhension de tels projets supranationaux et favoriser, j'ose l'espérer, l'adhésion à l'idée d'une Europe plus solidaire. C'est aussi une arme intéressante pour lutter contre les différentes formes de spéculation.

nous réjouissons de cette occasion, car elle nous permet de rappeler l'attachement du groupe RDSE aux enjeux européens, lequel passe par un engagement de tous les instants pour expliquer à nos concitoyens comment les institutions européennes contribuent à leur quotidien.

Elle met ainsi l'accent sur quatre points principaux : l'amélioration de l'efficacité des instruments de précaution ; la création d'un filet de sécurité autour du Fonds de résolution unique ; le renforcement et l'indépendance du mécanisme ; et, enfin, l'inscription d'une nouvelle règle de vote s'appliquant aux cas de restructuration. En tant qu'europhiles convaincus et, je l'espère, convaincants, nous sommes évidemment favorables à cette ratification qui, à nos yeux, permet de consolider les fondations du projet européen. Aujourd'hui, il semble nécessaire d'enrichir L'enjeu est d'ailleurs de taille, puisque l'un des objectifs sous-jacents de ce texte est la solidarité. Je rappelle que le MES dispose déjà de différents outils témoignant de l'esprit d'entraide qui caractérise l'Union européenne. Je pense ici à la possibilité pour les États membres en difficulté de se voir accorder des taux d'intérêt plus faibles, ou encore à la possibilité d'accorder des prêts aux banques privées, afin de maintenir, non seulement les systèmes financiers nationaux, mais surtout l'équilibre financier supranational. Si je m'attarde sur cet enjeu de société primordial qu'est la solidarité, mes chers collègues, c'est notamment parce que nous ne pouvons pas adopter des solutions inéquitables et qui excluent, dans cette période de crise sanitaire qui a indiscutablement fragilisé l'économie. Selon les estimations du programme de stabilité 2021-2027, la dette publique française ne diminuerait qu'à partir de 2027. C'est pourquoi j'estime que le renforcement du MES par l'instauration d'un nouveau filet de sécurité va dans le bon sens.

Quoi qu'il en soit, alors que l'Union européenne apparaît de plus en plus comme une tour de Babel pour certains, ou un Léviathan impuissant pour d'autres, il est fondamental que nous gardions confiance dans les solutions européennes, qui constituent et matérialisent un espace de compromis éclairé, gage de sécurité et de stabilité financières. Aussi, pour toutes ces raisons, le groupe RDSE est favorable à ce projet de loi et le votera à l'unanimité

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la crise de 2008, qui a atteint son paroxysme en Europe au début de l'été 2012, a révélé l'urgence d'une union bancaire.

le Conseil européen a décidé de doter l'Union européenne d'un mécanisme de surveillance bancaire, de modalités de résolution ordonnées des faillites bancaires et de filets de sécurité financiers. parallèle, le Mécanisme européen de stabilité a été créé par accord intergouvernemental pour gérer les problèmes de refinancement des dettes des États membres de la zone euro en temps de crise.

instaurées par les trois plans d'aide successifs dont le pays a bénéficié en 2010, 2012 et 2015, pour éviter la faillite, ce qui l'aurait contraint à sortir de la zone euro et à abandonner la monnaie unique.

État se vide d'une partie de sa jeunesse, à la recherche d'un meilleur avenir dans d'autres pays européens. Aujourd'hui, les dommages causés par la cure d'austérité appliquée à la Grèce en contrepartie des aides qui lui ont été accordées soulèvent la question de la responsabilité des institutions européennes.

preuve à la fois de solidarité et de souplesse pour mobiliser toutes leurs capacités financières communes et placer l'investissement au coeur de leurs politiques économiques de gestion et de sortie de crise. Le MES pourrait apparaître aujourd'hui

il est impensable que le Parlement européen, seul organe tirant sa légitimité de la volonté démocratique des citoyens européens, reste à l'écart des procédures. Quatrièmement, cette réforme est une occasion manquée de faire du MES un véritable « Trésor européen », car chaque pays ne reste responsable que de sa propre part de risque. de la zone euro viennent pourtant de démontrer, même si c'est de manière temporaire, qu'ils sont capables d'accepter un partage collectif des risques, en prévoyant une somme qui serait solidairement garantie par les pays. Dans une version idéale, les parlements nationaux émettraient la garantie destinée au fonds sans la relier à un pays ou à une crise spécifique.

constat que notre continent n'était plus une « jungle concurrentielle » et que les pays membres entendaient, ensemble, mieux protéger leurs citoyens en favorisant l'emploi et la formation. Nous pouvons toutes et tous nous féliciter de cette évolution nécessaire. le plan de relance historique adopté durant la crise sanitaire, doté de ressources propres, a posé les fondements de cette nouvelle politique. J'en profite pour saluer l'engagement de nos députés européens dans les négociations, lorsque beaucoup n'y croyaient pas.

nous voterons ce matin en faveur du projet de loi autorisant la ratification de l'accord modifiant le traité instituant le Mécanisme européen de stabilité. Cet accord, signé en début d'année par les dix-neuf États membres de la zone euro, introduit quatre un point majeur, il crée un filet de sécurité autour du Fonds de résolution unique. Il permettra au MES de prêter jusqu'à 68 milliards d'euros au Conseil de résolution unique, c'est-à-dire l'agence européenne chargée de la résolution des difficultés rencontrées par les établissements de crédit, afin de pallier, à titre exceptionnel, subsidiaire et temporaire, une éventuelle insuffisance des ressources du FRU. L'objectif est simple : faire en sorte que le contribuable ne soit pas celui qui vient au secours des banques en difficulté, comme ce fut le cas en 2008 et 2009.

Il renforce par ailleurs les compétences et l'indépendance du MES, en particulier concernant l'évaluation de la soutenabilité des dettes des pays de la zone euro et la négociation des réformes en cas de programme d'assistance financière. Il a enfin pour objet de simplifier la restructuration de l'endettement public d'un État, en réduisant le risque qu'un groupe minoritaire de créanciers s'y oppose dans l'espoir d'obtenir, par la suite, de meilleures conditions de remboursement. Le MES fournit une aide financière aux États membres qui connaissent, ou qui seraient susceptibles de connaître, de graves problèmes de financement. L'accord vient donc consolider un outil de gestion de crise, qui contribue à maintenir la stabilité financière de la zone euro. Cette mesure va dans le bon sens. Par ailleurs, la Commission européenne vient de lancer une consultation sur la révision des règles budgétaires au sein de l'Union, sujet au coeur de la future présidence française en 2022. Il s'agira de réduire la dette, tout en évitant d'entraver la croissance et de ralentir les investissements en faveur de la transition écologique.

Capus. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, on nous demande aujourd'hui d'autoriser la ratification d'un accord modifiant un traité intergouvernemental, et ce afin de renforcer une union économique et monétaire, elle-même établie par l'Union européenne. À n'en pas douter,

Au sein de la commission des finances, nous savons que l'emprunt commun européen consenti lors de la crise sanitaire aura un coût. Cette avancée historique découle d'une solidarité régionale dont nous pouvons nous enorgueillir. Toutefois, une dette doit être remboursée, même si elle est émise à plusieurs. Aussi, au-delà des ressources propres, nous avons besoin d'une stabilité économique, financière, monétaire et bancaire. Il m'est impossible, dans les quelques minutes qui me sont imparties, d'évoquer précisément les évolutions qui ont été négociées en vue de la révision de cet accord. J'aimerais toutefois revenir sur deux d'entre elles, qui me semblent essentielles pour l'avenir.

est à mettre en parallèle avec la place des États- par l'intermédiaire de leurs ministres des finances -, qui reste prépondérante dans les prises de décision. Cela fait partie du perfectionnement recherché dans un système qui n'a pas encore trouvé sa forme définitive. il crée le fameux filet de sécurité pour le Fonds de résolution unique. Cette précaution supplémentaire augmente la voilure du MES et des dispositifs qui l'entourent. de stabilité revisité est synonyme de solidarité, de stabilité et de fiabilité pour la zone euro. C'est la raison pour laquelle le groupe Les Indépendants votera en faveur de ce projet de loi de ratification.

le Mécanisme européen de stabilité a été créé pour faire face à une crise de la dette souveraine au sein de la zone euro, à l'instar de celle que nous avons connue à la suite de la crise financière de 2008. Elle avait conduit les chefs d'État et de gouvernement de la zone euro à décider, en 2010, la mise en place d'un dispositif européen pérenne, se substituant à des mécanismes temporaires, et de nature à garantir la stabilité financière en Europe. Les dirigeants européens avaient alors pris conscience de la nécessité de sortir d'une simple logique de sauvetage si nous voulions, à terme, parvenir à une stabilité économique et budgétaire durable.

Il permet ainsi aux pays de ladite zone de bénéficier d'un mécanisme permanent de gestion des crises à même de protéger les économies européennes contre les attaques spéculatives. Bénéficiant de capitaux propres fournis par les États membres de la zone euro selon une clé de contribution de contribution préétablie, le MES est autorisé à lever des fonds en émettant des instruments financiers, et en concluant des accords ou en négociant des arrangements financiers avec ses membres, des institutions financières ou d'autres tiers.

répondre présent pour faire face à une crise survenant dans un pays tiers et comment ces sommes seraient provisionnées.

Tel a été l'objet des travaux conduits en 2018 et 2019 pour réviser le traité de 2012 : ceux-ci ont abouti à la signature, les 27 janvier et 8 février 2021, d'un traité révisé, dont la ratification est soumise à l'accord des parlements nationaux.

davantage d'outils pour promouvoir la soutenabilité de la dette des États membres ; une participation plus active à la préparation aux crises ; un accès simplifié aux lignes de crédit de précaution du MES, afin d'empêcher l'aggravation de crises mineures ; un rôle plus important dans la conception et le suivi des futurs programmes d'assistance ; enfin, filet de sécurité pour le Fonds de résolution unique, pour renforcer le mécanisme de résolution des défaillances bancaires. Ce dernier point est essentiel : le filet de sécurité doit garantir que les États et, partant, les contribuables, ne seront pas mis à contribution en dernier ressort, en cas de défaillance d'une banque de la zone euro.

à charge pour ce dernier de rembourser ensuite le prêt, une hausse des contributions des établissements financiers et bancaires. C'est donc seulement dans le cas où tous ces verrous de sécurité se révélaient insuffisants que les États seraient mis à contribution. Le rapporteur de notre commission, dont je tiens à saluer la qualité du travail, a souligné l'importance de ce nouveau filet de sécurité, tout en mettant en exergue trois points de vigilance.

Le mécanisme de résolution unique est l'un des trois piliers de l'Union bancaire votée par le Parlement européen le 15 avril 2014, avec le mécanisme de supervision unique des banques européennes par la Banque centrale européenne et le système unique de garantie des dépôts, un fonds de

Il s'agissait en effet, après l'étape préalable et incontournable de la supervision commune, de veiller à ce que l'Union européenne, et non plus chaque État membre, soit en mesure de faire face financièrement et politiquement aux défaillances bancaires, sans que les contribuables soient mis à contribution. Le financement du mécanisme de résolution unique repose sur les banques elles-mêmes, à travers des contributions au Fonds de résolution unique qui, jusqu'en 2024, doivent permettre d'atteindre le niveau cible de 1 % du total des dépôts garantis, soit environ 75 milliards d'euros.

Je m'interroge : pourquoi ce changement ? Quelle est la raison impérieuse qui le justifie ? Quel est l'objectif de cette manoeuvre ? Mes chers collègues, doit-on considérer que notre présence, nos amendements, nos échanges sont à ce point inutiles que l'on peut nous imposer un calendrier à la dernière minute, sans nous en expliquer la cause réelle et sérieuse ? Ou considère-t-on que le texte de la commission des lois vaut loi sans même avoir été voté ? de nos débats, c'est un mépris pour nos collègues. J'espère, monsieur le président, qu'à défaut d'avoir été prévenus en temps voulu nous aurons au moins une explication sur ce changement d'horaire ! Acte

mesdames, messieurs les sénateurs, me voici devant vous pour vous présenter, au nom du Gouvernement, le onzième projet de loi sur la gestion de l'épidémie de covid-19. Comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire ici lors lors de l'examen des précédents textes sur le sujet, ce n'est pas avec enthousiasme que le Gouvernement présente un nouveau projet de loi permettant de prendre des mesures de freinage qui affectent la vie quotidienne de l'ensemble de nos compatriotes. Mais l'ampleur et la durée de la crise sanitaire exigent une mobilisation permanente des pouvoirs publics pour lutter contre ce virus toujours présent au quotidien, lequel a emporté la vie de près de 5 millions de personnes dans le monde, dont 117 000 dans notre pays. Néanmoins, nous pouvons prendre un instant pour nous retourner et mesurer le chemin parcouru depuis le début de la crise, ainsi que les progrès réalisés pour mieux gérer cette épidémie dans la durée, et limiter au mieux ses conséquences sanitaires et ses effets sur notre vie quotidienne. Ainsi, en métropole, la vague épidémique liée à la propagation du variant delta a pu être contenue, sans restriction généralisée de la circulation des personnes ou des rassemblements et en maintenant ouverts l'ensemble des établissements, et ce grâce au passe sanitaire et aux progrès significatifs de la campagne de vaccination. La mobilisation de tous et l'esprit de responsabilité de chacun ont permis d'atteindre des résultats tout à fait remarquables. À ce jour, plus de 51 millions de personnes ont reçu au moins une première dose. Bientôt, près de 50 millions de nos compatriotes auront un schéma vaccinal complet. C'est l'une des meilleures couvertures vaccinales d'Europe. Nous pouvons collectivement en être fiers, car c'est le fruit de la mobilisation de tous, notamment des collectivités territoriales que vous représentez et qui ont été au rendez-vous. En matière de vaccination, il ne faut relâcher nos efforts sous aucun prétexte. La campagne de rappel, lancée le 1septembre dernier, est à ce titre un rendez-vous crucial. Par ailleurs, nous amplifions les opérations d'« aller vers » pour progresser sur la vaccination de nos concitoyens éloignés du système de santé, en particulier des personnes les plus fragiles et les plus âgées. Néanmoins, à l'heure où je vous parle, nous sommes confrontés à un risque de rebond épidémique, à l'approche de la période hivernale, propice à une accélération de la circulation virale. Quasiment tous les pays européens sont confrontés à une hausse du nombre des cas, la situation étant inquiétante en Europe de l'Est. ministre déléguée ! Dans notre pays, on observe depuis quelques jours une tendance moins favorable et une reprise de la circulation épidémique. Sans évoquer à ce stade une cinquième vague, nous devons être particulièrement vigilants. Dans les prochains mois, nous devrons donc continuer à respecter certaines mesures barrières qui, bien qu'allégées par rapport aux phases les plus critiques de l'épidémie, demeurent indispensables. À cet égard, le Gouvernement lance une grande campagne d'information rappelant l'importance du respect des gestes barrières face au relâchement observé chez certains de nos concitoyens depuis plusieurs semaines. C'est particulièrement important alors que nous entrons dans une période de mise sous tension de notre système de santé du fait de la circulation simultanée de la covid-19, de la bronchiolite, de la grippe et de la gastro-entérite. Personne ne souhaite un nouvel emballement de l'épidémie, dont les conséquences humaines seraient à nouveau dramatiques et perturberaient encore fortement la vie de notre pays. Pour continuer à disposer d'outils permettant de protéger la population contre les phases les plus aiguës de propagation de l'épidémie, le projet de loi qui vous est soumis prévoit de proroger jusqu'au 31 juillet 2022 la validité du cadre juridique de l'état d'urgence sanitaire, fixée aujourd'hui au 31 décembre Je précise qu'il s'agit non pas de pouvoir activer pour une durée illimitée le régime de l'état d'urgence sanitaire pendant cette période, mais uniquement de maintenir les dispositions du code de la santé publique qui en fixent les règles, s'il apparaissait nécessaire de le déclarer. Un décret en conseil des ministres restera nécessaire à cette fin, et sa prorogation au-delà d'une durée d'un mois ne pourra être autorisée que par le Parlement. En Guyane, région confrontée à une circulation virale toujours inquiétante, l'état d'urgence sanitaire en vigueur sera prorogé jusqu'au 31 décembre.

que le Gouvernement peut, par décret pris après avis du conseil scientifique, décider d'y mettre un terme anticipé si la situation le permet. Le projet de loi proroge également jusqu'au 31 juillet 2022 le régime de gestion de la crise sanitaire, sur lequel repose actuellement la gestion de l'épidémie pour l'essentiel du territoire national. La prorogation de ce régime est la condition du maintien des mesures barrières dans les prochains mois. proroge également, jusqu'à la même échéance, la possibilité de mobiliser par voie réglementaire le passe sanitaire, outil qui a fait ses preuves, puisqu'il a permis de concilier le maintien de nombreuses activités avec une maîtrise de la circulation du virus. Les modalités de recours au passe sanitaire ont été précisées par l'Assemblée nationale. Sa mise en oeuvre sera justifiée par la circulation virale ou ses conséquences sur le système de santé, selon des indicateurs que le pouvoir exécutif devra prendre en compte, et ce sous le contrôle du juge administratif, comme c'est le cas depuis le début de la crise sanitaire. Pendant la période visée par ces prorogations, nous avons prévu un dispositif d'information du Parlement et la remise, d'ici la mi-février, d'un rapport qui présentera les mesures prises pour freiner l'épidémie et qui justifiera, le cas échéant, la nécessité de les maintenir pour la période restante. Ce dispositif d'information du Parlement a été enrichi par l'Assemblée nationale, qui a apporté des précisions sur la production d'indicateurs sanitaires et la remise d'un second rapport d'ici la mi-mai et de rapports d'étape mensuels. La remise d'un rapport au mois de février constituera une clause de revoyure, qui s'ajoutera à l'ensemble des initiatives prises depuis le début de la crise, afin d'assurer l'information du Parlement sur la gestion de l'épidémie. Je pense en particulier aux dossiers transmis chaque semaine aux présidents des deux assemblées et aux réunions du comité de liaison organisées régulièrement par le Premier ministre. Par ailleurs, le texte améliore plusieurs outils importants pour garantir l'efficacité de la gestion de l'épidémie dans les prochains mois. Ainsi, nous proposons de renforcer la lutte contre la fraude au passe sanitaire en aggravant les sanctions encourues en cas d'établissement, de proposition ou d'utilisation d'un faux passe sanitaire, et en permettant à l'assurance maladie de contrôler les certificats de contre-indication à la vaccination. qui concerne l'obligation vaccinale pour les soignants, le texte prévoit d'améliorer son contrôle et son effectivité, notamment en autorisant les écoles de santé à contrôler son respect par les étudiants en santé, et et en ouvrant la possibilité pour les établissements employeurs d'accéder directement au statut vaccinal des professionnels soumis à cette obligation, sous réserve, toutefois, qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale Par ailleurs, nous proposons de prolonger jusqu'à la fin du mois de juillet les systèmes d'information SI-DEP et Contact Covid qui sont, comme vous le savez, des outils absolument indispensables pour suivre la situation sanitaire et « casser » les chaînes de contamination. Sur ce sujet, le texte a été complété par une disposition permettant aux directeurs d'établissement scolaire d'accéder aux informations relatives au statut virologique et vaccinal des élèves. Cette disposition vise à donner à ces directeurs d'établissement les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la campagne de vaccination et de dépistage dont ils ont la charge, ainsi qu'à l'application des protocoles sanitaires dans les écoles, les collèges et les lycées. La situation actuelle, reposant sur des déclarations parentales, ne permet pas, en effet, de fiabiliser ni d'affiner les mesures prises et de limiter ainsi les fermetures de classes dans l'intérêt des élèves. Enfin, le texte proroge un nombre ciblé de mesures d'accompagnement, qui permettront de faire face en tant que de besoin aux conséquences de la crise sanitaire, notamment en en matière d'activité partielle ou de fonctionnement des organes délibérants des collectivités territoriales. Vous l'aurez compris, le projet de loi qui vous est soumis ne bouleverse pas l'économie générale de la gestion de la crise sanitaire, mais il conforte les différents outils dont nous disposons pour y faire face. Dans un contexte toujours incertain, et face au risque de voir émerger de nouveaux variants, plus transmissibles ou plus pathogènes, une grande vigilance s'impose face à un virus avec lequel nous savons d'ores et déjà que nous devrons vivre au moins jusqu'à l'été prochain. C'est bien ce souci d'anticipation et cette vigilance qui ont guidé le Gouvernement dans l'élaboration du texte qui vous est présenté. Ce texte, votre commission des lois l'a très largement modifié, en ramenant tout d'abord au 28 février 2022 l'échéance des différents régimes qu'il prévoit. Ainsi que l'a indiqué le ministre des solidarités et de la santé lors de son audition, le Gouvernement est néanmoins déterminé à retenir comme horizon le mois de juillet 2022. En effet, nous savons très bien dès à présent qu'il nous faudra vivre avec le virus au moins jusqu'à l'été. La période hivernale sera en tout état de cause propice à une aggravation de la situation. Le rapport prévu pour la mi-février, je l'ai dit, permettra au Parlement de disposer d'une clause de revoyure. Il pourra bien entendu donner lieu à un débat en commission ou en séance, en présence du Gouvernement.

Les remplacer par de nouvelles dispositions créerait de la complexité et de l'insécurité, alors que le cadre existant a été éprouvé. Le Gouvernement ne juge pas non plus opportun d'inscrire dans la loi un taux précis de vaccination pour la mise en oeuvre de tout ou partie des mesures, notamment du L'inscription d'une valeur spécifique directement dans la loi ne manquerait pas de rigidifier la gestion de la crise. Ainsi que l'a souligné le conseil scientifique dans un récent avis,

D'autres modifications ont été apportées aux dispositions consacrées aux mesures d'accompagnement de la gestion de crise, afin de tirer les conséquences des évolutions apportées aux premiers articles du texte. Vous l'aurez compris, mesdames, messieurs les sénateurs, nous avons des désaccords sur la solution à proposer et l'horizon à retenir pour gérer la suite de l'épidémie de covid-19. Sans épuiser l'ensemble des divergences, ... C'est sûr ! ... le Gouvernement a déposé plusieurs amendements

proportionnées à l'évolution de la situation, afin de protéger la santé de nos concitoyens dans les meilleures conditions. Mes chers

c'est le onzième projet de loi dont nous sommes saisis. Chaque fois que nous l'avons été, nous avons répondu présents : nous avons assumé nos responsabilités et donné au Gouvernement et aux autorités sanitaires les outils, les moyens, les instruments dont ils avaient besoin

Ce n'est pas nous, madame la ministre, qui changeons de pied lorsque nous disons que nous ne voulons pas vous donner les pleins pouvoirs pour lutter contre la covid-19 jusqu'au mois de juillet prochain. C'est vous qui en avez changé

point de masques, point de gel hydroalcoolique, point de tests de dépistage, point de vaccins, point de télétravail, point de respect des gestes sanitaires et des mesures de distanciation sociale. Bref, nous n'avions rien pour faire face à l'intrusion de ce virus sur la scène nationale, alors même qu'il avait été détecté dès le mois de décembre.

de cette nouvelle étape, qui a débuté à l'Assemblée nationale la semaine dernière, il convenait d'adapter nos outils à la réalité sanitaire, laquelle a a heureusement évolué dans le bon sens, tant du point de vue de la vaccination que du rythme des contaminations. Nous sommes face à une situation nouvelle, qui justifiait d'ailleurs qu'on en débatte. Si nous vous avions laissé, comme vous le demandiez, les pleins pouvoirs en matière sanitaire jusqu'au 31 décembre, nous n'en débattrions pas aujourd'hui. Et il est d'autant plus nécessaire d'en débattre que, les choses ayant changé, nous pouvons ajuster nos instruments. L'idée toute simple que je vous propose de retenir est la suivante :

de faire un premier test puis, après une semaine, d'en faire un second. Pourquoi traiteriez-vous différemment les enfants ? Et puis, ces informations médicales, que va-t-on en faire ? Nous pensons que ce n'est pas raisonnable. Si encore

en oeuvre de l'obligation vaccinale a été globalement réussie. On peut estimer à près de 95 % la proportion des personnels des établissements sanitaires et médico-sociaux désormais engagés dans une démarche vaccinale contre la covid-19. Si les quelque 8 000 suspensions et 3 000 démissions liées à un refus vaccinal ont pu perturber le fonctionnement de certains établissements, elles ne doivent pas occulter l'esprit de responsabilité dont a fait preuve l'immense majorité des soignants. Comme l'a souligné le ministre devant notre commission, près des deux tiers des personnes suspendues ont finalement été réintégrées après s'être conformées à l'obligation vaccinale. Par contraste, la situation en outre-mer, tout particulièrement dans les Antilles et en Guyane, reste un sujet de préoccupation. Dans ces territoires, l'obligation vaccinale

Nous comprenons le dilemme auquel font face les autorités sanitaires dans ces territoires : faire respecter les lois de la République, tout en préservant les capacités de fonctionnement des hôpitaux ultramarins déjà sous tension. Le ministre a annoncé l'ouverture d'une médiation en Martinique pour surmonter ces difficultés. Sachez que la commission des affaires sociales du Sénat sera particulièrement attentive aux résultats de cette médiation pour rendre l'obligation vaccinale pleinement effective en outre-mer. Le projet de loi que nous examinons n'entend pas rouvrir le débat sur l'obligation vaccinale des professionnels au contact des personnes vulnérables, que le Parlement a tranché l'été dernier. L'article 3 se contente de simplifier les modalités de contrôle du respect de cette obligation, afin d'alléger, notamment, la charge de travail pesant sur les agences régionales de santé.

propres aux établissements ou par la complexité du contrôle à réaliser. Par ailleurs, s'agissant des sanctions pénales en cas d'usage de faux justificatifs vaccinaux, nous avons rétabli les peines introduites dans la loi du 5 août dernier, tout en réintégrant l'établissement de faux justificatifs de vaccination dans le champ des actes réprimés. Concernant les dispositions relatives au droit du travail, l'article 5 prévoit de prolonger jusqu'au 31 juillet 2022 plusieurs mesures exceptionnelles relatives au dispositif d'activité partielle. Ce terme nous a semblé bien trop lointain,

S'agissant, plus particulièrement, du complément employeur aux indemnités journalières versées par l'assurance maladie, le Gouvernement serait habilité à adapter ou à compléter par ordonnance des mesures prises par décret sur le fondement d'un dispositif permettant de déroger aux conditions de versement de cette indemnité en cas de crise sanitaire. demande est surprenante, puisque ces mesures sont déjà prorogées par le présent projet de loi. Pour ce qui concerne l'activité partielle de longue durée, pourquoi demander une habilitation aussi large si la mesure envisagée n'est que ponctuelle ?